tout rachat de capital d'une entreprise délégataire de service public conduisant à un franchissement du seuil de 25 % de détention des droits de vote au sein de ladite entreprise. Dans la période de crise sanitaire que nous vivons, l'action des collectivités territoriales doit être essentiellement tournée vers les mesures sanitaires visant à protéger la population et vers les mesures économiques et sociales visant à faire face aux conséquences Aussi, les opérations économiques conduisant à des changements majeurs dans l'organisation des délégations de service public, telles que le rachat de Suez par Veolia, ne conduiraient qu'à complexifier inutilement le travail des collectivités locales, en remettant en cause l'équilibre de services à la population. Le Gouvernement ayant mis en avant, sans succès, son opposition à ce projet, il pourrait, grâce à cet amendement, pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire, différer celui-ci afin de ne pas affecter les capacités d'action des élus locaux, dont l'attention pourrait être portée ailleurs.

ont besoin de s'adresser à des entreprises qui sont en concurrence les unes avec les autres pour pouvoir maîtriser les coûts des marchés qu'elles contractent avec leurs concessionnaires.

l'intrusion de l'État dans l'activité des entreprises est limitée par un texte fondamental, l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirme le principe du droit de propriété en même temps qu'il en énonce les limites. En effet, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'y a pas de principe sans limites, et il faut que les droits soient combinés entre eux pour pouvoir faire naître la réalité

excessives. Je profite aussi de cette occasion pour préciser ce que l'État et le Gouvernement font déjà depuis plusieurs années pour contrôler les opérations portant atteinte à certaines des entreprises stratégiques de notre territoire

L'Assemblée nationale a largement adopté, dans une récente loi de finances rectificative, une enveloppe de 20 milliards d'euros pour donner les moyens à l'État d'investir dans les sociétés menacées. Enfin, et ce n'est pas le moindre des arguments, le fonds Lac d'argent de la banque publique d'investissement, que

statuer ... Ce texte contient de nombreuses dispositions qui tirent les conséquences de la situation très particulière dans laquelle nous nous trouvons, y compris d'un point de vue économique. En réalité, j'entends, par vos explications procédurales, que vous êtes en désaccord sur le fond.

Il est donc hors de question de retirer cet amendement, malgré les éléments de procédure qui ont été rappelés par M. le secrétaire d'État. J'espère que nous réunirons une majorité au sein de cette assemblée pour défendre les intérêts de nos concitoyens.

faire l'objet d'un débat plus approfondi. Il y a urgence sanitaire, mais il y a aussi urgence économique. Il aurait été intéressant d'aller au bout de la réflexion à partir de cet amendement.

par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

que les conseillers prud'homaux soient autorisés à disposer chacun de deux pouvoirs, afin de limiter le nombre de ceux qui se réuniront. Pour mémoire, les élections respectives des présidents et vice-présidents des conseils prud'homaux, sections et chambres se tiennent chaque année au mois de janvier. La parole

Ces règles doivent en effet être assouplies afin de tenir compte des places disponibles dans les différents établissements.

ayant un besoin temporaire particulier ou auprès d'organismes non agréés, mais qui satisfont aux conditions de l'agrément. Cette dérogation et les mises à disposition qui en découlent prendront fin, en tout état de cause,

dont la moyenne d'âge est assez élevée, devant prendre des mesures de précaution qui peuvent les empêcher de prêter main-forte aux associations. Il est donc important pour ces dernières de pouvoir bénéficier de ce service civique.

d'État a fait un effort pour nous expliquer les intentions du Gouvernement, mais il n'a pas non plus été très précis. Actuellement, un certain nombre d'organismes agréés peuvent accueillir des jeunes qui bénéficient d'un contrat au titre du service civique, ce qui est très

ou d'autres organismes agréés. J'insiste sur cet adjectif, car il permet d'éviter toute forme d'abus dans l'utilisation de cette procédure extrêmement utile pour des jeunes qui souhaitent s'engager, au service de la société, dans des organismes à but non lucratif ou des établissements publics.

que représente ce service pour les jeunes qui ont décidé de s'y engager.

les organismes qui pourraient en bénéficier. Il s'agit des organismes d'accueil agréés qui ont été ajoutés par la loi du 17 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, des personnes morales de droit public français agréées, des organismes sans but lucratif de droit français agréés et, enfin, des organismes agréés ou qui satisfont aux conditions de l'agrément s'ils ne l'ont pas déjà. Une solution pourrait consister à inscrire directement

il est impératif d'insister sur les singularités de l'outre-mer afin de prendre en compte une situation épidémique ultramarine parfois différente de celle de l'Hexagone. De ce point de vue, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite une attention particulière, ses ressortissants qui souhaiteraient le rejoindre sont dans l'obligation de transiter par le territoire canadien. Ce transit constitue un risque élevé au regard de l'augmentation du niveau d'alerte au Canada. Or les passagers arrivant à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont actuellement plus soumis à une mesure de quarantaine. Certes, la préfecture préconise fortement aux personnes concernées de respecter une période d'autoconfinement de sept jours, mais un tel dispositif nous paraît insuffisant- il doit être renforcé et rendu coercitif. Il s'agit d'une demande expresse de notre collègue de Saint-Pierre-et-Miquelon Stéphane Artano, qui souligne que cette carence est la source d'une vive inquiétude dans l'archipel. Cet amendement tend à imposer à tous ceux qui entreraient sur le territoire de l'archipel

Nous n'avons pas à ériger au niveau législatif, pour la seule visite de touristes étrangers à Saint-Pierre-et-Miquelon, cette règle qui permettrait de mettre en oeuvre une quatorzaine à l'arrivée sur le territoire de cette

a repris les dispositions précédentes sur les mises en quatorzaine, et elles sont bien évidemment applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces mises en quatorzaine doivent toutefois être prononcées dans le cadre prévu par la loi. Ainsi, à l'entrée sur le territoire, elles ne peuvent être prescrites qu'à l'égard des personnes ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection. Ce classement est fixé par arrêté, et, au vu de sa situation sanitaire, le Canada n'y figure pas à ce jour. Pour autant, cette liste est appelée à être actualisée en fonction de l'évolution de la situation.

par avion à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent en tout état de cause présenter le résultat négatif d'un examen de dépistage de moins de soixante-douze heures pour pouvoir embarquer. J'ajoute que les tests par RT-PCR ne sont plus les seuls examens présentant une fiabilité suffisante pour la détection du covid-19. Les travaux sont déjà bien avancés pour nous

localement au préfet, en concertation avec les forces économiques et sociales et la communauté médicale, de prendre toutes les mesures pour protéger la santé de la population et réduire la circulation du virus. C'est ce qu'a fait le

et sociaux provoqués par la crise sanitaire et les mesures mises en oeuvre pour la combattre. Par conséquent, adopter une disposition absolument générale-

l'avis du Gouvernement ?

l'Assemblée nationale a introduit l'obligation de présenter un projet de loi de ratification au Parlement dans un délai d'un mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Le Parlement pourra donc contrôler le contenu de ces ordonnances et leur conformité à l'habilitation initiale lors de l'exercice de ratification. À cette occasion, il

M. le rapporteur. Une loi qui prévoit que la durée de son application est déterminée dans une certaine limite de temps par un décret n'est pas inconstitutionnelle. De la même façon, si une ordonnance le fait, elle ne sera pas contraire à nos règles fondamentales. Puisque vous avez rappelé, ce dont je me réjouis, que j'ai été secrétaire général de la présidence de la République, sachez que je n'ai aucune raison de le cacher- j'en suis au contraire très fier ! Et je dois dire que le Président Jacques Chirac, que j'ai servi pendant huit ans

Le présent amendement a pour objet de mettre en place des dispositions semblables au profit des particuliers. Il s'agit de les protéger eux aussi de l'encours d'intérêts, de pénalités ou de toute mesure financière, action, sanction ou voie d'exécution forcée pour retard

pour des personnes qui travaillent dans des entreprises qui seront fermées de manière administrative ou dont l'activité dépend de ces entreprises. Il n'y a pas de raison de protéger les entreprises et pas les salariés. Quel est l'avis

C'est une question qui a une dimension sociale que tout le monde perçoit- je n'y reviens pas -, mais qui a aussi une dimension juridique. En échange de son loyer, l'entrepreneur

pour simplifier, on pourrait dire que l'entrepreneur n'en a plus pour son argent. Ce n'est pas la faute du propriétaire, ce n'est la faute de personne, c'est la faute d'une situation qui fait que le bien ne peut pas être exploité dans les conditions pour lesquelles le bail a été conclu.

certain nombre de difficultés d'application liées tant à la détermination de son champ d'application qu'à des questions d'indemnisation des propriétaires. D'autre part, elle ignore- permettez-moi de le rappeler -les nombreuses mesures qui ont été prises pour soutenir les personnes en difficulté dans le paiement de leur loyer.

la période précédente a montré l'engagement des banques pour trouver les aménagements nécessaires avec leurs clients en difficulté. Soyez convaincus que nous continuerons d'être attentifs

taper sur Action Logement ... Je veux également évoquer tous les coups de canif que vous avez mis dans le contrat concernant les aides au logement pour les particuliers,

répété de manière ferme.

De nombreux compatriotes ne peuvent se déplacer dans les postes consulaires compétents pour la délivrance de ces documents pour y effectuer les démarches nécessaires. Il s'agit particulièrement de nos compatriotes résidant à l'étranger âgés, handicapés ou confinés. Les services numériques dédiés à ces procédures ne fonctionnent pas toujours dans certains pays. Par ailleurs, les tournées consulaires sont limitées par la crise. Dans certains pays, l'obtention d'un visa est conditionnée à une date d'expiration du passeport intervenant au moins six mois avant la date de séjour. Certains États estampillent les visas de séjour temporaire directement sur le passeport, ce qui place le titulaire d'un passeport périmé en situation irrégulière au regard des services de l'immigration. Nous proposons donc que ces titres soient prorogés pour une durée de six mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Quel est l'avis de la commission ? Je remercie

au pire de la crise, 50 000 Français résidant à l'étranger n'avaient pas la possibilité d'aller récupérer leur passeport. La situation continue à être difficile.

se fait particulièrement prégnante. Un certain nombre de collègues ne veulent pas entendre parler de la mise en place du RSA jeune. Il faut pourtant s'interroger : dans un pays comme le nôtre, avec les sommes que le Gouvernement est capable de débloquer pour venir en aide aux entreprises en difficulté, mais également à leurs salariés,

sociales et alimentaires, mais aussi psychiques, parce qu'ils étaient cloîtrés chez eux, dans des chambres universitaires, très loin de leur famille

Nous savons tous que, sous le régime de la V République, le rapport de force entre l'exécutif et le législatif s'est inversé en défaveur du Parlement. J'ose dire que, chaque fois que nous demandons un rapport au Gouvernement, au lieu faiblesse du législatif par rapport à l'exécutif. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur tous les amendements tendant, pour

Cette crise a conduit l'État à apporter un soutien opérationnel et financier significatif aux opérateurs de l'alimentaire, tout en confortant son rôle de coordination, afin d'aider les acteurs à faire face à l'urgence et à la hausse des besoins. Deux premiers plans de soutien à l'aide alimentaire, dotés de 94 millions d'euros, ont été déployés dès le mois d'avril afin de soutenir les associations confrontées à des difficultés logistiques, mais aussi pour mettre en place une aide d'urgence alimentaire au profit des foyers les plus en difficulté, dispositif qui a été complémentaire de la distribution de chèques services à hauteur de 50 millions d'euros à destination des personnes sans abri. Ces décisions s'inscrivent dans l'ensemble des mesures sociales d'urgence prises afin d'aider les plus précaires face à la crise, dans des proportions jamais connues dans l'histoire de notre pays. Au total, elles ont représenté plus de 3 milliards d'euros de soutien direct aux personnes précaires. Le Gouvernement a par ailleurs renforcé son rôle de coordination des différents acteurs et dispositifs dès le mois de mars, en permettant la continuité des distributions grâce au réseau préfectoral. Ainsi, la circulaire du 2 juillet 2020 demande aux préfets de créer une instance de coordination opérationnelle pérenne au niveau départemental. Le Gouvernement a également installé le comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire au début du mois Face aux conséquences de la crise, le plan France Relance comporte une mesure de 100 millions d'euros pour soutenir les associations de lutte contre la pauvreté. Les associations engagées dans la lutte contre la précarité alimentaire sont particulièrement ciblées dans ce dispositif. Par ailleurs, conformément aux engagements du Président de la République, les montants des fonds européens consacrés à l'aide alimentaire ont été sanctuarisés, voire augmentés. Les commandes réalisées grâce au FEAD sont en train d'arriver et celles qui ont été effectuées au moyen des crédits React-UE sont en cours d'élaboration. En ce qui concerne le renforcement des mesures sanitaires, rassurez-vous, le décret d'application et l'attestation ouvriront une dérogation pour les personnes vulnérables, les travailleurs sociaux et les bénévoles travaillant la nuit, notamment dans le cadre de maraudes sociales. Enfin, pour être complet,

d'appeler l'attention du Gouvernement sur la situation de ces personnes et de lui demander de faire en sorte que tout soit mis en oeuvre pour les protéger au maximum.

Par ailleurs, le Gouvernement a procédé, cet été, à l'expédition par La Poste de 53 millions de masques lavables pour les foyers modestes. Cette opération est en cours de renouvellement. Ce seront à nouveau plus de 50 millions de masques qui vont arriver dans les boîtes aux lettres d'ici à la mi-novembre, une une troisième opération étant d'ores et déjà prévue. Pour les personnes sans abri, près de 52 millions de masques jetables ont été expédiés dans les préfectures à la fin du mois d'août, pour une distribution les CCAS et les associations. Cet envoi va être reproduit,

une « confusion absolue entre les notions de " confinement sanitaire " et d'" isolement psychiatrique " », aboutissant à des privations de liberté injustifiées et illégales selon le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire ne doit pas être l'occasion d'un retour à de telles dérives.

des mesures mises en place par ces établissements de santé dans le cadre d'une cellule de crise nationale, qui rassemble les différents acteurs. Consécutif à une décision du Conseil constitutionnel du 19 juin dernier,

précise les dispositions du code de la santé permettant de mieux encadrer juridiquement le recours aux pratiques d'isolement et de contention en psychiatrie. Elles entreront en vigueur à compter du 1 janvier prochain. Les dispositions proposées par le Gouvernement répondent aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, en posant justement des durées maximales et en définissant les modalités d'encadrement et de contrôle des mesures d'isolement et de contention prises dans le cas des soins sans consentement. Elles visent également à accroître les garanties en matière de droits des patients, en renforçant la motivation des décisions médicales, mais également leur traçabilité tant au sein du dossier médical du patient qu'au sein du registre de suivi de ces mesures. En réalité, par ces nouvelles dispositions, la France se met en conformité avec les conventions internationales, en développant un meilleur contrôle et en renforçant la politique active de réduction de ces pratiques déjà engagée, sans méconnaître pour autant la réalité de la situation difficile à laquelle sont confrontés les professionnels et les nécessités cliniques qu'impose la prise en charge des patients. Le Gouvernement est défavorable à votre demande de rapport.

pendant la durée d'application de l'état d'urgence sanitaire, afin de pouvoir assurer leur disponibilité pour des missions de réserve sanitaire, militaire, de police ou de sécurité civile, dans un contexte de forte tension opérationnelle pour l'ensemble de ces services ». Le présent amendement a pour objet d'étendre ce dispositif aux agents contractuels de la fonction publique. La commission a regretté de ne pas y avoir pensé toute seule ... C'est dire si elle se réjouit de cet amendement, sur lequel elle a émis un avis favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Favorable.

à Mme Jocelyne Guidez. La date des élections départementales et régionales est, en théorie, fixée aux 14 et 21 mars 2021, mais le Gouvernement souhaite les reporter pour des motifs sanitaires. Dans ces conditions, et en l'absence de nouvelle date, les départements et les régions se trouvent privés d'outils de communication par l'article L. 52-1 du code électoral, qui dispose que, dans les six mois précédant un scrutin, aucune communication institutionnelle inédite ne peut être faite. Cette situation est préjudiciable à l'intérêt général. Par exemple, les entreprises en difficulté, les commerçants, les TPE et indépendants ne peuvent pas avoir accès à l'information sur les dispositifs d'aide d'urgence. De même, les demandeurs d'emploi ne peuvent être informés, par une campagne de communication, des nouveaux dispositifs d'aide et de formation mis en place à leur intention. Cette situation peut avoir des conséquences économiques et sociales dramatiques pour les intéressés.

de laisser en déshérence tant d'entreprises en difficulté économique et sociale sans les informer de ce que les aides leur permettent

que ces collectivités ne peuvent pas mener de « campagne de promotion publicitaire » de leurs réalisations ou de leur gestion. Il s'agit là d'une mesure essentielle- vous me rejoindrez sur ce point, madame la sénatrice -pour assurer l'égalité entre les candidats et ne pas privilégier les sortants en leur offrant les moyens de la collectivité pour leur campagne. M. le rapporteur le rapporteur ne semble pas en accord avec l'interprétation du Gouvernement. Pourtant, cet article n'empêche pas les collectivités d'informer les entreprises ou les particuliers sur les dispositifs ouverts, à condition que cette information ne donne pas lieu à une autopromotion, et ce sous le contrôle du juge de l'élection.

de toute la législation qui vise à mettre en situation équitable les candidats à une élection. Le président d'un exécutif local dispose d'une capacité de communication qui est aussi une capacité financière

de limiter la communication autorisée par les collectivités locales pour qu'elle ne vire pas à la propagande électorale. Il ne faut pas confondre l'information, qui est tout à fait légitime jusqu'au dernier jour du mandat,

plus ou moins les moyens de leur collectivité pour mener des opérations de communication électorale. Ce n'est pas possible ! J'appelle donc votre attention sur ce point.

et c'est normal ! Le code électoral et la législation sur le financement des campagnes ont vocation non à empêcher les élus d'exercer leur mandat jusqu'à leur terme, mais à mettre les candidats en situation équitable. Je comprends que le rapporteur soit quelque peu

ce n'est pas simple, d'autant plus que, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, l'État, comme l'ensemble des collectivités territoriales, s'implique fortement aux côtés de tous les partenaires.

dès lors qu'elles ne valorisent pas leur action. J'appelle l'attention du rapporteur et du président de la commission des lois sur ce point

et il me semble que ce ne serait pas envoyer un bon message au juge administratif que de l'appeler, par le biais de cet amendement, à une tolérance ou à une pondération dans les jugements qu'il prononcera sur les élections municipales.

très fermement opposés à ces deux amendements.

Sur l'initiative de notre collègue Éric Kerrouche, un dispositif avait été proposé, mais on nous avait opposé à l'époque, ce qui était factuellement exact, que le temps était très court et qu'il serait sans doute complexe de mener cette opération à bien pour le second tour du scrutin.

correspondance, qui nous paraissent plus adaptées et permettent sa sécurisation, sans faire dépendre la possibilité de cette modalité d'exercice du droit de suffrage de l'état d'urgence sanitaire, dont on sait qu'il peut être un jour prolongé, le lendemain abandonné, le surlendemain repris. Quel est

associer publiquement l'ensemble des parties prenantes, il a été décidé de confier à M. Jean-Louis Debré une mission pour étudier les conditions dans lesquelles pourraient se tenir les scrutins

Les conclusions de cette mission devraient être rendues d'ici à trois semaines. Je vous propose d'attendre qu'elles soient remises avant de procéder à une évolution

pour achever cette formalité qui est plus que substantielle. Par conséquent, dans le cadre des mesures liées à l'état d'urgence sanitaire et, surtout, au confinement, cet amendement vise à repousser au 8 janvier la date de dépôt des comptes de campagne.

l'avis du Gouvernement ?

Dans une démocratie, on ne change pas le calendrier des élections, quelles qu'elles soient, sans un motif d'intérêt général extrêmement puissant. Le seul motif pour lequel on pourrait reporter les élections locales prévues au mois de mars prochain, c'est naturellement un motif de sécurité sanitaire, si le déroulement de la campagne puis le déroulement du scrutin devaient avoir une incidence négative sur la santé publique en exposant nos concitoyens, en premier lieu les candidats, à des risques de contamination. Il faut donc d'abord s'attaquer au problème de la sécurité de la campagne électorale, et à la sécurité du scrutin avant d'envisager un report. Partir de l'idée que la seule question posée serait celle du report revient à restreindre

Faudrait-il commencer par se poser la question de réviser l'article 6 de la Constitution, qui prévoit la date de la fin du mandat présidentiel, avant de s'interroger sur notre capacité

de différer des élections pour des motifs de convenance politique, il vous faut démontrer d'abord, non pas que vous vous êtes interrogé sur la date d'un scrutin, mais que, conscient de votre

nous ne pourrons pas attendre au-delà du 31 décembre prochain pour savoir si les élections doivent se tenir ou pas.

les conclusions de la mission menée par Jean-Louis Debré pour pouvoir, en toute transparence, collectivement, parce que nous aurons établi les conditions de sécurité

cette intention du Gouvernement et nous l'avons concrétisée en introduisant dans notre texte un assouplissement du régime des procurations. Ces deux éléments permettront de sécuriser le scrutin. Si vous le souhaitez, vous pouvez fort bien ne pas attendre

Les deux dispositifs proposés, qui ont fait l'objet de discussions en commission des lois, posent une question de fond et de forme. Sur le fond, des considérations constitutionnelles sur les injonctions du Gouvernement nous invitent à exprimer une certaine prudence. Sur la forme, cet amendement tend à exiger du Gouvernement ce qu'il a en réalité déjà annoncé, à savoir une décision à la fin de l'année sur la tenue des scrutins de mars 2021, 2021, à l'issue de la mission confiée à Jean-Louis Debré, qui consulte aujourd'hui et travaille à l'émergence d'un consensus sur la question afin que les élections, ainsi que la campagne qui les précède, puissent se tenir dans les meilleures conditions.

car ces frais ne sont pas différents en période de covid et en période de sécurité sanitaire.

que les frais d'incidents bancaires soient plafonnés pour les publics les plus vulnérables. Vous connaissez le dispositif : plafonnement à 25 euros par mois de tous les frais d'incidents ; plafonnement à 20 euros par mois et à 200 euros par an des frais d'incidents pour les bénéficiaires de l'offre spécifique que les banques doivent proposer à leurs clients en situation de fragilité ; augmentation de 30 du nombre de bénéficiaires de cette offre spécifique. En 2020, le ministre de l'économie et des finances a signé un décret pour mieux encadrer encore l'identification des publics fragiles. Je n'entre pas dans le détail. Le principe du plafonnement des frais d'incidents bancaires et l'ensemble des mesures que nous avons prises sur ce sujet ont été consignés dans une charte qui a été homologuée par décret du ministre de l'économie et des finances. nous avons resserré le suivi de cette question. L'Observatoire de l'inclusion bancaire a été chargé de relever chaque trimestre les données à ce sujet, au lieu de deux fois par an Il analysera notamment la façon dont les banques détectent la fragilité et le nombre de personnes concernées. Sur la base du prochain bilan de l'Observatoire, nous serons prêts à enrichir le dispositif actuel, en concertation, évidemment, avec les parlementaires qui travaillent activement sur ce sujet. La parole est à Mme Nathalie Goulet,

parce qu'elles craignent d'être contaminées en se rendant dans un établissement hospitalier. Cette crainte, nous dit-on, pourrait perdurer après la fin du confinement, le virus n'ayant pas disparu, comme le prouvent d'ailleurs les décisions de reconfinement qui ont été prises par le Gouvernement. Pendant toute la période qui a suivi la fin du premier confinement, un certain nombre de femmes peuvent ne pas avoir été rassurées à l'idée de se rendre dans des services hospitaliers ou avoir vu leur mouvement entravé. C'est donc sur

comporte des inconvénients beaucoup plus importants que pendant la période précédente. Tous ces éléments combinés me font penser qu'il ne faut modifier les échéances prévues dans la loi

nous explique ce qu'il met en oeuvre pour assurer le respect des droits des femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse avant d'envisager une telle mesure. La commission, comme elle l'avait fait lors des deux précédents examens du même

le rétablissement par voie réglementaire des adaptations pour l'IVG médicamenteuse pour préserver le droit à l'avortement pendant cette phase d'urgence sanitaire, le recours à la téléconsultation, à la vidéoconsultation pour la prise des médicaments- le rapporteur l'évoquait -, ainsi que la facilitation du retrait des médicaments nécessaires en pharmacie, ou encore l'extension de deux semaines de la période pendant laquelle l'IVG médicamenteuse peut être pratiquée, soit jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse. L'ensemble de ces mesures est en cours d'examen dans le cadre nouveau du confinement tel qu'il a été établi par le Président de la République, puis précisé par le Premier ministre hier. Nous sommes en train d'évaluer quelles dispositions doivent être réactivées,

visant à renforcer le droit à l'avortement, à l'Assemblée nationale, le 8 octobre dernier, le Gouvernement s'est engagé- et a saisi le Comité consultatif national d'éthique à cette fin -à étudier la perspective d'étendre de façon pérenne les délais impartis pour pratiquer l'IVG hors période de crise sanitaire.

cette configuration de vie très particulière a provoqué une explosion des violences intrafamiliales. Le ministre de l'intérieur avait constaté, au bout de dix jours de confinement, 32 % d'augmentation des signalements dans les zones gendarmerie, 36 % pour la préfecture de police de Paris.

à l'interdiction de se déplacer, et donc au couvre-feu ou à ce qui en tient lieu désormais, et ne peuvent pas être maintenues en confinement dans le même domicile que l'auteur des violences. Si l'éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d'hébergement doit leur être attribué.

La commission a déjà permis l'adoption d'un amendement de même nature pour ce qui concerne les quarantaines. Il s'agit là aussi de mettre à l'abri une personne menacée de violences conjugales ou ayant subi de telles violences pendant la période du confinement, même si celle-ci est plus souple que la précédente. La commission a émis un avis favorable.

l'avis de la commission ? Tout d'abord, pendant cette période de confinement, l'accès aux plages n'est pas interdit ; c'est très important. important. Ensuite, il est vrai que nous avons voulu, au moment de la sortie du premier confinement, faciliter l'accès aux activités nautiques. C'était d'autant plus possible et souhaitable que nous arrivions à la période de l'été et que la vitesse de circulation du virus était extrêmement faible.

par des décisions du Gouvernement sont suffisantes et qu'il ne faut pas aller au-delà. L'avis de

Pour autant, les activités nautiques, je me permets de le préciser, restent interdites. La parole

contre ce projet de loi, pour plusieurs raisons que ma collègue Cécile Cukierman a eu l'occasion de rappeler lors de la discussion générale. Bien évidemment, nous ne méconnaissons pas les efforts qui ont été réalisés par la commission des lois, notamment par son rapporteur. Il n'en demeure Il n'en demeure pas moins que ce texte donne toujours trop de pouvoirs à l'exécutif, et pendant beaucoup trop longtemps, en abaissant le rôle du Parlement. Je pense sincèrement qu'il s'agit d'une démission démocratique. Or nos propositions pour redonner au Parlement la place et le rôle qui doivent être les siens, particulièrement dans une situation de crise, ont été rejetées. Nous en prenons acte.

du travail. Nous rappelons une nouvelle fois que c'est une façon de mettre à l'écart le Parlement, d'autant que la Constitution n'est pas respectée, celle-ci exigeant une ratification expresse des ordonnances, ce qui est,

et inquiet que nous portions sur ce projet de loi, en raison de la négation du rôle du Parlement, mais aussi de l'absence de tout un pan de nécessaires dispositions dans le domaine social dans cette période. Incontestablement, et nous avions déposé des amendements en commission, nos regards ont convergé avec la majorité de la commission, puis

Des progrès très importants ont donc été réalisés et nous en sommes satisfaits. Pour autant, le Sénat a systématiquement refusé

de tout faire pour ne pas revivre un épisode aussi dramatique que celui du printemps dernier. Il faut agir rapidement et avec force. C'est dans ces circonstances que la prorogation de l'état d'urgence sanitaire paraît indispensable, tout comme il paraît nécessaire d'habiliter le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance durant cette période, mais toujours avec le sens de l'urgence et de l'intérêt général. Comme je le disais lors du débat sur la déclaration du Gouvernement, un vote favorable ne signifie ni une unanimité irréfléchie ni un blanc-seing. mes collègues du groupe RDSE et moi-même nous réjouissons du travail effectué en vue de la réduction du nombre des habilitations accordées au Gouvernement. Le Parlement ne doit pas être écarté de toute décision durant cette crise et nous demandons à être associés aux orientations que le Gouvernement souhaite impulser. La gravité de la période ne saurait suffire à justifier une atteinte si excessive aux principes régissant le fonctionnement démocratique de notre nation. Car la démocratie doit pouvoir se poursuivre, au niveau national comme au niveau local. En ce sens, le groupe RDSE se félicite de l'adoption de l'amendement déposé par notre président, Jean-Claude Requier, assouplissant les règles de quorum applicables aux organes délibérants des collectivités territoriales. Il paraissait impératif d'accompagner nos collectivités territoriales dans leur action quotidienne. Nous pensons aussi à nos compatriotes d'outre-mer, qui subissent cette crise dans des conditions particulières. Il faudra donc veiller à ce qu'ils reçoivent notre soutien tout au long de cet épisode, comme nous avons souhaité le faire en particulier pour nos concitoyens de Saint-Pierre-et-Miquelon.

ses territoires. Au regard de tous ces éléments, le groupe RDSE votera en faveur de ce texte. Comme j'ai déjà pu le souligner, notre position est commandée par l'intérêt général. Elle est une position de raison, un soutien de responsabilité face aux événements. Toutefois, ce vote ne nous empêchera pas de rester vigilants. Le Parlement devra toujours demeurer en mesure d'assumer l'une de ses principales fonctions : celle de contrôler l'action du Gouvernement. La parole

intéressante, mais ardue. En tout cas, elles ont permis de tester la bienveillance des sénatrices et des sénateurs. Le Sénat s'est efforcé,

permettez-moi de « zoomer » sur ce sujet. Les masques transparents ont fait l'objet de certifications très rapides grâce à la mobilisation du secrétariat d'État chargé du dossier,

Je n'allongerai pas les débats outre mesure, mes chers collègues. Plusieurs points n'apparaissaient pas irréconciliables au commencement. Je pense à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, à laquelle nous avons en majorité consenti dans cette assemblée. Je pense également aux mesures d'urgence économique et sociale. Si un désaccord a pu se poser quant à la méthode, si une certaine méfiance, que nous ne partageons pas, a pu s'exprimer sur ces bancs, nous nous accordons tous, je le crois, sur le caractère indispensable de ces mesures. Un certain nombre d'amendements, y compris du Gouvernement, sont d'ailleurs venus depuis hier soir renforcer les dispositifs proposés pour tirer les conséquences, très difficiles, de cette crise. Certaines réserves importantes demeurent dans les modalités de gestion de la crise : je pense à la faculté de mettre en oeuvre, à l'issue de l'état d'urgence un régime transitoire conférant une certaine agilité et de nature à favoriser une sortie anticipée de celui-ci. Je pense également à l'allongement très modeste que prévoit ce texte pour la mise en oeuvre des systèmes d'information,

raisonnable ou pas de voter après les décisions, si la gestion de la crise sanitaire était pertinente ou non et si finalement la société française était suffisamment résiliente pour résister aux conséquences des mesures qui étaient prises. C'était oui ou non, blanc ou noir. En cette fin de matinée, nous avons à nous positionner sur un texte

a demandé que le Parlement soit en situation d'être saisi, au plus tard le 8 décembre, et qu'il se prononce une mesure de prorogation du reconfinement. Cela change tout ! Sur cette base, le groupe Union Centriste est clairement favorable au projet

je ne ferai pas le reproche au Président de la République de vouloir faire une mauvaise utilisation des cinq mois et demi d'état d'urgence, mais nous nous d'urgence, mais nous nous mettons à accepter une situation d'affaissement de notre démocratie qui, dans un autre contexte politique, nous placerait dans une situation impossible. Ne créons pas ce genre de précédent.

qu'est l'état d'urgence sanitaire soit la solution adéquate. Ce régime est en effet bien trop attentatoire aux libertés individuelles et publiques. Des mesures doivent évidemment être prises, mais elles se doivent d'être raisonnées et proportionnées, et le Gouvernement ne peut exclure la participation du Parlement dans le processus décisionnel. Bien entendu, nous saluons le travail de la commission des lois, de son rapporteur et des sénateurs ici présents pour améliorer considérablement le projet de loi qui était présenté par le Gouvernement et pour en faire un objet, non pas désirable, mais acceptable. Toutefois, je me permets de mentionner, pour ceux qui pourraient avoir besoin d'un petit rappel, que les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire, malgré les modifications qui ont été apportées, permettent de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes et des véhicules, de réglementer l'accès aux moyens de transport, d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile, d'ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine de personnes susceptibles d'être infectées, d'ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, d'ordonner la fermeture provisoire et de réglementer l'ouverture de plusieurs catégories d'établissements et de commerces recevant du public, de limiter ou d'interdire les rassemblements, d'ordonner la réquisition de toute personne nécessaire à la lutte contre les catastrophes sanitaires, de prendre des mesures temporaires de contrôle des prix, etc. La liste de ce que permet cet état

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur

dans l'incapacité de faire appel à des fonctionnaires des États membres en raison de doutes sur les potentiels conflits d'intérêts. Les pouvoirs publics ont besoin de restaurer toute la validité de l'expertise des scientifiques. Pour cela, il faut un système clair

de Marco. L'indépendance de la recherche passe également par la transparence des liens d'intérêt avec des entreprises et autres personnes morales de droit privé.

On constate également que le mode actuel de recrutement des professeurs ou des directeurs de recherche marginalise les économistes ne s'inscrivant pas dans le cadre de la pensée économique dominante. le maintien d'un minimum de pluralisme intellectuel dans l'enseignement supérieur et la recherche en économie est remis en cause. Pourtant, la tradition hétérodoxe française, riche et diverse, a toujours participé au rayonnement international de la France. Aujourd'hui, face notamment, mais pas seulement, à l'incapacité pour la théorie dominante d'envisager la possibilité ou la prévention de crises financières, les économistes hétérodoxes réclament une réévaluation majeure de la pensée et des politiques macroéconomiques. La disparition du pluralisme en économie se traduit également par un appauvrissement de l'enseignement de l'économie à l'université. L'offre universitaire en économie est de moins en moins diversifiée. Elle ne répond plus aux attentes des étudiants, qui réclament de manière récurrente un enseignement ancré sur l'analyse du monde réel et des enjeux économiques et sociaux actuels. L'hégémonie d'une pensée dominante en économie se traduit de fait aussi par un tarissement des financements de la recherche sur certains territoires, avec une concentration des flux financiers vers les universités et laboratoires Cela conduit à Cela conduit à de fortes inégalités territoriales, particulièrement pénalisantes pour les universités et les laboratoires de recherche concernés, qui sont généralement constitués de petites et de moyennes structures.

sens. Voilà qui permettrait de préserver la diversité des écoles de pensée en économie et de soutenir institutionnellement le pluralisme de la recherche et de l'enseignement. Notre débat démocratique s'en trouverait également grandement enrichi. Ne l'oublions pas, à l'origine, cette science s'appelait « économie politique

mais également dans le monde, où des positions dites « hétérodoxes » peuvent ne pas recevoir toute l'attention qu'elles méritent. Mais l'avis

Quand une science n'arrive pas à décrire le réel, c'est qu'il faut peut-être se poser des questions et envisager de revenir au débat contradictoire entre les disciplines.

l'adoption de cette loi et des ordonnances du 22 septembre 2017, les dispositions du code du travail sur la durée du travail et les congés sont organisées selon le triptyque suivant : d'abord, l'ordre public, auquel aucun accord ne peut déroger, sauf dans un sens plus favorable aux salariés,

au contexte et au fonctionnement propre des passerelles permises entre les activités de recherche privée et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche publique. L'amendement n° 116, présenté

de recherche dans le double objectif de remettre la négociation collective au centre du dispositif et d'éviter de faire reposer des charges excessives sur les entreprises.

à une prise de congé qui entraînerait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Ensuite, la condition d'ancienneté supplétive serait d'un an seulement

afin de coller davantage au régime de congé pour création ou reprise d'entreprise. Quel est l'avis de la commission

telle réforme pose problème. Le cas spécifique des primes d'encadrement doctoral n'est plus pris en compte. En conséquence, les avis de la commission de la recherche et du conseil académique sont supprimés. Les versements des primes seront donc soumis à la totale discrétion des chefs d'établissement. On peut aussi s'interroger sur la généralisation d'un tel système de récompenses au mérite.

que du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quel est

Ensuite, la répartition des compétences entre le conseil d'administration et le chef d'établissement me paraît pertinente : le conseil arrête les principes et le chef d'établissement est responsable de l'attribution. Enfin, l'article précise clairement que les primes d'intéressement ne sauraient se substituer au régime indemnitaire. Cela constitue une garantie très attendue dans les établissements. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Cela n'est pas pertinent. Le combat pour l'égalité doit reposer non pas sur l'attribution de primes- cela pourrait laisser penser que le régime indemnitaire de base est inégalitaire -, mais plutôt sur les conditions dans lesquelles les chercheuses et les enseignantes peuvent mener leur carrière. Je rappelle également que l'axe 3 de l'accord du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique prévoit déjà de supprimer les situations d'écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.